La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Ainsi, il ancre dans la loi le principe de la différenciation territoriale en offrant aux collectivités certaines attributions afin d'y parvenir. Dans cette perspective, il apparaît essentiel que les services de l'État soient associés à ce processus, afin, d'une part, de faciliter sa bonne réalisation, et, d'autre part, d'assister au mieux les collectivités territoriales dans leur effort de différenciation. Il s'agit de dire non pas que les collectivités devraient être limitées en raison de l'action étatique des services déconcentrés, mais que ces services facilitent la réalisation de la différenciation territoriale et les initiatives locales de nos collectivités ainsi que les expérimentations qu'elles peuvent mener. Il s'agirait ainsi d'inaugurer une nouvelle culture administrative de partenariat renforcé et de travail partagé.

puisque les services déconcentrés de l'État ont déjà pour mission de favoriser la réalisation des initiatives locales, y compris en matière de différenciation territoriale, dans le cadre de la mission de conseil et d'accompagnement que les préfets

qui pointait déjà les limites actuelles du droit en matière de différenciation territoriale pour les outre-mer. Bien qu'inscrit dans la Constitution,

un prérequis : la nécessité de l'actualisation régulière, de la simplification et de l'adéquation législative du droit à la différenciation pour nos territoires d'outre-mer. Quel est l'avis de la commission ? Chère collègue,

Toutefois, la rédaction que nous proposons a vocation à s'appliquer à tous les territoires qui, aujourd'hui, ne disposent pas de ce droit à la différenciation. Or les territoires ultramarins bénéficient déjà de dispositions particulières. Vous évoquez la mise en oeuvre des dispositions de la loi. Je me permettrai d'inviter

encadre de manière peut-être excessive les pouvoirs du Parlement. En effet, le législateur doit demeurer libre de légiférer, lorsque la situation le justifie, pour simplifier ou adapter le droit spécifiquement

l'amendement n° 390 est-il maintenu ? Madame la ministre, sachez que, lors de l'élaboration de ce rapport, quasiment tous les exécutifs des différents territoires ont été auditionnés

collectivités d'outre-mer. Dès lors, on peut s'étonner que l'étude d'impact annexée à ce projet de loi précise que les mesures de l'article 1 ne s'appliquent pas en outre-mer.

Madame la ministre, nous devons aller plus loin dans la décentralisation et la simplification, pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées. La décentralisation de la compétence médico-sociale est loin d'être parfaite et l'entrelacement des compétences entre l'État, l'assurance maladie et les départements rend la gouvernance illisible et cloisonnée et la coordination de l'accompagnement difficile à mettre en oeuvre. C'est pourquoi je pense que nous devons décentraliser l'ensemble de la compétence médico-sociale à l'échelon s'agit d'améliorer la coordination et la prise en charge des personnes handicapées, âgées et dépendantes, dans la perspective de la réforme du grand âge. Je suis favorable à un transfert du budget soins- autrement dit, des Ehpad -aux conseils départementaux, qui sont déjà responsables des budgets hébergement et dépendance. De la même manière, dans le secteur de l'aide sociale, je pense que nous devons transférer aux départements le budget

d'aide et de soins à domicile qui regroupent SSIAD et SAAD pour plus de coordination. Concernant l'accompagnement des personnes handicapées en établissement, les foyers de vie sont placés sous la responsabilité des départements, alors que leur médicalisation relève du budget de l'État. Aussi, je pense que nous devons aller vers un partage plus homogène des blocs de compétences et faire du département l'autorité unique d'organisation et de tarification des établissements et services qui relèvent du champ médico-social.

À défaut, ces propositions pourraient ne jamais obtenir de réponse, comme l'expérience l'a malheureusement démontré, notamment pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse. Cet amendement vise donc à prévoir un mécanisme à deux niveaux

après censure du Conseil constitutionnel, permet cependant à la collectivité de Corse de demander à être habilitée par le législateur, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île. ans plus tard, force est de constater que cet article est totalement inopérant alors même que les spécificités de la Corse ont été reconnues depuis lors dans l'arsenal législatif, notamment dans la loi Montagne. Madame la ministre, vous le savez mieux que moi, la quasi-totalité des demandes adressées par la collectivité de Corse au Gouvernement sont restées sans réponse, preuve du caractère purement cosmétique de cet article et de l'indifférence des gouvernements successifs. Le présent amendement, conformément à l'esprit de ce projet de loi qui entend redonner la parole aux territoires, vise à rendre opérationnels les pouvoirs d'expérimentation et d'adaptation dévolus à la collectivité de Corse. Je me réjouis que mon collègue Panunzi s'aligne sur les demandes de la collectivité de Corse. C'est la preuve, madame la ministre, qu'il existe une convergence politique sur cette question, que vous ne pouvez ignorer.

nous avons demandé un pouvoir de différenciation concernant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.

les jours d'ouverture et de fermeture. Cette demande est restée lettre morte. Nous n'avons jamais eu de réponse malgré toutes nos demandes. Nous attendons aujourd'hui que le Gouvernement nous fasse un signe

Les propositions de modification d'ordre réglementaire peuvent également faire l'objet d'une transmission afin de permettre au Parlement de suivre ces demandes au titre de son pouvoir de contrôle de l'action du Gouvernement.

il appelait de ses voeux à « repenser en profondeur l'interaction entre l'État et les collectivités » afin de redonner « aux territoires les moyens d'agir dans une responsabilité partagée ».

ouvrait ainsi la voie à la reconnaissance d'espaces de vie différenciés sur le territoire national. Cette révision constitutionnelle a disparu du calendrier présidentiel au mois d'août 2019.

ne permettra pas d'améliorer significativement les interactions entre l'État et les collectivités, une telle amélioration étant pourtant indispensable à une réconciliation entre les citoyens et leur administration et à un retour de la confiance.

entre la France et l'Allemagne. Ce traité prévoit que les deux États s'engagent à doter les collectivités territoriales des territoires frontaliers

adopté

des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement » des départements. La Collectivité européenne d'Alsace

J'ai, comme chacun d'entre nous, beaucoup de respect et de considération pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mais une telle disposition lui permettrait

L'avis est absolument semblable à celui de la commission. Monsieur Jacquin, je suis étonnée que vous demandiez que des départements, même frontaliers, puissent signer des engagements internationaux.

: le président de ces collectivités peut demander à représenter l'État pour un accord particulier. Le dialogue international se fait bien évidemment d'État

C'est un véritable casse-tête pour les élus, qui ne savent pas quelle règle doit être appliquée. Cela entraîne une insécurité juridique des décisions prises par les collectivités lorsqu'une loi est respectée et que l'autre ne l'est pas.

sur l'article. L'article 2 porte sur l'extension du pouvoir réglementaire local, dans le cadre de concertations territoriales entre les collectivités et l'État. C'est bien dans ce cadre que l'enseignement facultatif des langues régionales est conduit dans notre pays.

La situation des langues régionales, affaiblie par la dernière censure du Conseil constitutionnel, aurait dû trouver une réponse dans un texte dont l'un des piliers est la différenciation.

Mme Laurence Cohen. La commission a modifié l'article 2 afin de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales, notamment le règlement départemental d'aide sociale. Cette modification peut paraître anodine au premier abord, mais, si chaque département élabore son propre règlement pour l'attribution des aides sociales, nous franchirons un pas supplémentaire vers la segmentation et la division de l'unité nationale.

d'ignorer l'actualité juridique : les tribunaux administratifs ont toujours annulé les règlements départementaux qui ont tenté de limiter ou de réduire l'accès au RSA. Par ailleurs, autoriser le transfert des reliquats du budget de la prestation de compensation du handicap vers le budget général des départements reviendrait automatiquement à réduire les dépenses départementales en faveur de la compensation du handicap. Ces deux dispositions nous semblent extrêmement régressives. C'est pourquoi nous en demandons la suppression. L'amendement

par mois. Gabriel Garcia Marquez écrivait : « J'ai appris qu'un homme n'a le droit d'en regarder un autre de haut que pour l'aider à se relever. » Notre amendement s'inscrit dans cet esprit. La parole est à M. Guy Benarroche,

à l'égard des bénéficiaires des dispositifs sociaux. La plupart des études convergent pour montrer que les bénéficiaires de minima sociaux veulent retrouver un emploi

des modifications qui touchent aux droits des plus vulnérables de nos concitoyens ! Nous ne pouvons pas accepter

droit, on cherche à traquer les quelques économies qu'une personne aurait pu réaliser durant sa vie avant de perdre son emploi

Je le dis très tranquillement à nos deux rapporteurs : si on voulait décrédibiliser l'idée de différenciation territoriale, on ne s'y prendrait pas

Cela nous semble contraire à l'esprit de l'ensemble des dispositions relatives aux missions et aux statuts des CCAS et CIAS. À nos yeux, si un centre intercommunal venait à être dissous, ses attributions devraient de plein droit être restituées aux communes ou à leurs CCAS, et non être exercées directement par l'EPCI. L'objet de cet amendement est de repenser la répartition des attributions du centre dissous au bénéfice des seules communes.

de déterminer librement les représentants à associer au sein de la Commission consultative des services publics locaux sans restreindre la participation aux seules associations locales. Cet amendement vise à ouvrir plus largement

Deuxièmement, il est proposé de supprimer la disposition relative à la détermination de la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser) par délibération du conseil régional.

qui est susceptible d'aller à l'encontre de la récente décision du Conseil constitutionnel et qui a été introduite dans le texte sans avoir attendu les conclusions de la mission parlementaire demandée par le Premier ministre.

qui permettent d'éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Le Ceser a su s'adapter à sa mission de relais de l'opinion publique en tenant compte des nouveaux appétits démocratiques de nos concitoyens.

que les Ceser soient dorénavant composés non plus par décret en Conseil d'État, avec une mise en oeuvre confiée au préfet de région, mais par les conseils régionaux, dans les trois mois suivant leur renouvellement.

Ce changement risque d'apporter confusion et doutes quant à l'impartialité de la parole des Ceser. La défiance des Français envers nos institutions risque de n'en être que plus grande. Dans un contexte où les niveaux d'abstention sont de plus en plus importants et inquiétants, il est

peuvent, par l'adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des voeux sur la mise en oeuvre de cette convention afin qu'elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d'enseignement, permettant d'assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale.

ministre. Je ne suis pas une spécialiste des langues régionales, et ce n'est pas mon ministère qui gère ce dossier.

matière et que les produits phytosanitaires sont considérés comme nocifs pour la santé humaine, rien ne permet aujourd'hui à un maire d'agir pour la préservation de la santé environnementale de ses administrés. Pourquoi ne pas écouter ces maires, que vous connaissez tous, quand ils souhaitent limiter les épandages de pesticides trop près des écoles ? Pourquoi ne pas les écouter quand ils perçoivent un danger en matière de pollution du sol ou de contamination des eaux ?

de la santé. Un maire ne peut pas intervenir dans ce champ, puisque la décision du ministre de la santé annule toute initiative particulière.

Vous proposez d'ajouter aux pouvoirs de police municipale des cas spécifiques de réglementation des produits phytopharmaceutiques. Conformément aux exigences de la réglementation européenne, la police spéciale de la mise sur le marché de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est confiée à l'État par la loi. Le code rural et de la pêche maritime encadre fortement la mise en oeuvre de cette police spéciale, qui s'appuie sur des évaluations scientifiques approfondies. Les produits phytopharmaceutiques font l'objet d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il appartient ensuite au ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé de la santé, de l'environnement et de la consommation de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits. Puis, le préfet de département est chargé de fixer les distances minimales d'utilisation des produits à proximité des lieux accueillant des personnes. Le Conseil d'État a précisé dans son arrêt du 31 décembre 2020, c'est-à-dire très récemment, que le maire ne peut légalement user de ses pouvoirs de police générale pour édicter une réglementation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu'il appartient aux seules autorités de l'État de prendre. Pour autant, le projet de loi Climat et résilience, dans son article 49 D, renforce le rôle du maire, au titre de sa compétence aménagement et urbanisme, en prévoyant qu'il peut définir des zones de transition entre zones urbanisées et agricoles au travers de son Chacun est ainsi conforté, si je puis dire, dans ses compétences, que le Gouvernement n'entend pas modifier. J'émets donc un avis défavorable sur cet

Un maire peut n'avoir aucune connaissance des stratégies structurelles dans l'installation d'un certain nombre de sources d'énergie comme les éoliennes. Un maire peut très bien n'avoir aucune connaissance des dangers supposés des éoliennes. Un maire peut très bien n'avoir aucune connaissance des dangers des pesticides. Nous sommes bien d'accord ! Néanmoins, y a-t-il moins de possibilités pour un maire de connaître la dangerosité de l'épandage de pesticides à cinq mètres d'une école, alors qu'il a peut-être des retours d'un certain nombre

: La parole est à M. Ludovic Haye. Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales concourt aujourd'hui à deux principes structurants du droit des collectivités territoriales : la libre administration des collectivités territoriales et la différenciation. L'article 2 du projet de loi, largement enrichi par Mme la rapporteure Françoise Gatel, vise à une extension du pouvoir réglementaire locale dans plusieurs domaines. Il prévoit notamment la fixation par une délibération du conseil municipal du régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux.

la mission de dresser la liste des constructions exonérées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Vous m'avez entendu, les conseils municipaux auront la mission mission - quelle compétence ou quelle responsabilité ont-ils dans ce cas ? - de dresser la liste des constructions exonérées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Je le répète, parce que cela paraît énorme. Cette disposition est actuellement fixée par décret en Conseil d'État.

Nous ne pouvons pas prendre le risque d'un débordement s'agissant de l'exonération de normes encadrant les constructions. Ce sont ces normes qui ont permis d'atteindre de nouveaux standards environnementaux.

de vous donner un exemple. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, que certains connaissent, il y a un élevage de moutons de prés salés.

Monsieur Benarroche, votre amendement vise à revenir sur les modifications du code de l'urbanisme introduites par la commission. Premièrement, le fait de conditionner la prise en compte des observations du représentant de l'État à l'entrée en vigueur d'un document d'urbanisme permet, je crois, de vérifier la prise en compte réelle des enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols ou de répartition équilibrée des logements. Leur mauvaise prise en compte expose les communes et les porteurs de projet à une certaine insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle je pense que la sécurisation et le conseil, par des experts, auprès des collectivités territoriales permettent

il n'est pas souhaitable de confier à la collectivité le soin de déterminer les critères pour soumettre ou non un projet à autorisation d'urbanisme sans l'encadrer. Le fait de disposer d'une procédure de délivrance d'autorisations d'urbanisme identique sur tout le territoire permet donc une sécurité juridique pour les pétitionnaires. Cela facilite le montage et la sortie des projets. Il n'est pas souhaitable de le remettre en cause, en période de relance. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable

Au sein des zones d'aide à finalité régionale (ZAFR), la Commission européenne autorise les autorités françaises à octroyer des aides spécifiques. Ces aides contribuent au développement de ces zones en soutenant plus particulièrement les investissements initiaux des grandes entreprises et des PME et la création d'emplois liés à ces investissements. Afin de une plus forte cohérence de ces actions de soutien aux entreprises et une meilleure prise en compte des dynamiques territoriales, il apparaît opportun que les ZAFR soient définies

environnement ; elles en décident souverainement. D'un autre côté, les aides qui sont d'origine européenne voient leurs conditions d'attribution décidées un décret pris en Conseil d'État. Tout cela n'est pas très cohérent

d'octroyer, dans les territoires vulnérables, des aides aux entreprises en dérogeant au droit européen de la concurrence. Il s'agit d'un instrument privilégié pour atteindre les objectifs fixés en matière de cohésion territoriale la réduction des écarts de développement. Vous proposez que les régions soient les seules autorités à en définir la cartographie. Je suis évidemment convaincue du rôle des conseils régionaux, qui détiennent, comme vous l'avez rappelé, la compétence

cette méthode, qui permet de concilier la défense d'une position claire et lisible par la France et la concertation avec les collectivités régionales. En effet, ces AFR sont

ruraux des mesures fiscales et sociales. Au regard des responsabilités dévolues aux régions en matière économique et d'égalité des territoires, il est proposé, en déclinaison des SRDEII et

mais de ménager un minimum nécessaire avant tout destiné aux touristes et aux excursionnistes à vélo, ce qui relève d'une forme de standard national de service public. Il est donc normal que le seuil minimal reste fixé par le règlement national en vigueur.

En effet, le niveau minimum de performance énergétique est un élément essentiel pour apprécier la décence d'un logement. Néanmoins, à niveau de performance énergétique égal, l'habitabilité d'un logement sera objectivement différente selon qu'il est situé en plaine ou en montagne.

d'un élément concret de renforcement du pouvoir réglementaire des collectivités et de leurs groupements au bénéfice de la transition écologique. L'amendement

devient l'affaire de tous et si on laisse les collectivités territoriales prendre leur part. Les élus locaux connaissent bien leur territoire, ses spécificités, ainsi que les acteurs sociaux et économiques. Leur donner la possibilité d'aller plus loin dans le progrès écologique est un levier puissant, porteur d'avancées significatives.

de rénovation énergétique impliquant différentes dispositions coercitives à l'égard des bailleurs au travers de la caractérisation de l'indécence d'un logement pour raisons énergétiques. Celles-ci ont été fixées directement dans la loi de manière à la fois volontaire et mesurée, afin de ne pas déséquilibrer le marché immobilier et la location, tout en tenant compte des capacités de financement des maîtres d'ouvrage. Nous avons eu un débat assez long sur le sujet

le cadre réglementaire qui a été défini donne la possibilité aux intercommunalités ou à une commune de décliner à l'échelle du territoire des politiques encore plus ambitieuses de rénovation énergétique de l'habitat